adopté sous les réserves d’usage. J’informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi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 L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux

monsieur le ministre,

Or il est aujourd’hui parfois détourné, ce qui entraîne un gel excessif des projets, y compris dans des secteurs où les enjeux du logement, des énergies renouvelables et de la réindustrialisation sont cruciaux. De plus, un dispositif

Le sursis à statuer ZAN est un outil très important pour les maires en ce qu’il leur permet d’éviter que leur enveloppe foncière pour la période 2021 2031 ne soit complètement mangée avant qu’ils n’aient pu modifier leurs documents d’urbanisme.

en va de même pour les sources de financement dont elles pourraient bénéficier pour mettre en œuvre leurs projets de sobriété foncière. Comme nous l’avons évoqué hier, lors de la discussion générale,

dans la mise en œuvre de la politique de sobriété foncière. Cela vaut à la fois pour l’ingénierie et le financement. Dans le prolongement du « porter à connaissance » renforcé que nous avons prévu en commission,

pour valoriser des projets faiblement artificialisants dans une approche incitative, territorialisée et coordonnée. Ce bonus malus incitera à comparer plus systématiquement des projets, à concevoir différemment les opérations et à mieux intégrer la préservation des sols dans les politiques d’aménagement. Ce dispositif pourra servir également de point d’appui à la réforme de la fiscalité

La lutte contre l’artificialisation doit être pensée non pas en silo, mais comme faisant partie du mouvement de transition écologique. Parfois, artificialiser un peu plus sera,, bon pour l’environnement – je ne suis pas certain que tout le monde comprenne cette subtilité… Nous sommes donc favorables à cet amendement, qui va tout à fait dans le sens de la différenciation territoriale que nous défendons. Là où l’on trouve des projets vertueux pour l’environnement, il faut faciliter leur réalisation et donc céder un peu plus de foncier dans le cadre de la territorialisation. Quel est l’avis

Cet amendement vise donc à établir un mécanisme incitatif à la renaturation, permettant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’obtenir un droit à construire

Convenez que c’est quelque peu paradoxal… Compte tenu de coûts très élevés, un certain nombre de programmes d’accompagnement ont été mis en place. Il est indispensable que les EPCI, lorsqu’ils souhaitent se substituer aux propriétaires

La requalification des bâtiments agricoles, lorsqu’ils sont amiantés, est un défi. Comme nous le disons collectivement ici, l’objectif est de ne plus avoir de friches et de bâtiments qui seront, demain, des verrues et qui empêcheront tout aménagement et toute activité.

Les collectivités qui le souhaitent pourront ainsi s’emparer d’un outil de diagnostic complémentaire pour fonder leurs choix urbanistiques sur des paramètres pédologiques et privilégier l’artificialisation là où les sols sont de mauvaise qualité et où les performances agronomiques sont moindres ou déjà altérées. En effet, si de nombreux élus locaux font part de certaines difficultés à mettre en œuvre le ZAN, d’autres sont déjà bien engagés dans une démarche de ménagement du territoire. Je remercie les rapporteurs de l’avis favorable qu’ils ont bien voulu donner à cette expérimentation ambitieuse et je me réjouis de l’amendement identique déposé par le rapporteur pour avis Daniel Gueret. Nous sommes convaincus que les collectivités sauront se saisir de cet outil pour adapter l’aménagement du territoire aux contraintes climatiques et préserver nos sols avant même la transposition de la future directive européenne sur les sols. La France dispose d’un véritable leadership écologique sur la question des sols, grâce aux travaux menés par l’Institut national de recherche pour permettent d’inventer notre adaptation aux enjeux climatiques. Cette expertise offre la possibilité de poser les jalons d’une future politique nationale des sols. L’expérimentation proposée par cet amendement

Il est en effet scientifiquement regrettable qu’aucune distinction ne soit faite entre l’artificialisation d’un sol à haut potentiel agronomique et celle d’un sol plus pauvre ou aux fonctionnalités déjà altérées. Je me rends compte cependant que cette évolution est de nature à remettre en cause toutes nos habitudes urbanistiques. Une obligation qui s’imposerait à toutes les collectivités me paraît, à ce stade, très prématurée. Cependant, impulser cette évolution sous la forme d’une expérimentation me semble une démarche intéressante, qui permettra aux collectivités volontaires de favoriser des approches plus qualitatives en intégrant la qualité de leurs sols dans leurs documents d’urbanisme. Il s’agit par ailleurs d’un moyen d’anticiper concrètement les évolutions législatives en cours au niveau européen. C’est la raison pour laquelle je vous propose d’adopter cet amendement : cela offrirait aux collectivités du bloc communal qui le souhaitent d’expérimenter, en amont de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme, la réalisation d’un diagnostic relatif à la qualité et à la santé des sols du ressort territorial couvert par le document d’urbanisme. Quel est l’avis de la commission ? Je veux tout

et ne dédouane en aucun cas les collectivités qui souhaiteraient s’en emparer de leurs obligations au titre de la réglementation relative à la lutte contre l’artificialisation. Les retours

Deuxièmement, les modalités de l’objectif sont instables – il y a beaucoup trop de textes – et divergent d’un département à l’autre. En outre,

les élus qui seront à la tête de nos communes en 2044 ne seront vraisemblablement pas les mêmes

Je reprendrai un élément avancé hier par notre groupe lors de la discussion générale concernant l’insécurité juridique que fait planer la contractualisation évoquée sans enveloppe nationale contenant le nombre d’hectares possiblement ouverts à la consommation des Enaf. Sur quels critères se détermineront les préfets et les élus ? Légitimement, ces derniers considéreront que les projets qu’ils nourrissent dans leur territoire nécessitent une consommation d’Enaf. Qui pourrait

des objectifs qui étaient fixés initialement ! Je le dis en toute sincérité : quelle urgence y avait il à déposer ce texte plutôt que de nous accorder un peu plus de temps pour travailler conjointement sur les objectifs et sur les outils ? Quelle urgence y avait il à déposer ce texte avant d’avoir le retour ferme et définitif de la mission d’information sur laquelle nous travaillons pour faire le point sur les problématiques de financement ? Et le groupe de suivi ? On y

Il faut donc faire confiance aux élus, mais lesquels ? Dans un grand pays démocratique et moderne, l’État fixe des objectifs. Il considère qu’il faut lutter contre le changement climatique, et derrière le ZAN, on retrouve les enjeux majeurs d’adaptation au changement climatique et de lutte contre les inondations ; il estime qu’il faut

Dans ce cadre, l’élu clé est effectivement le conseiller régional, puisque nous avons confié la planification aux régions. Or vous fragilisez ici

qui ont déjà fait l’effort de s’inscrire dans une première trajectoire ambitieuse à l’horizon de 2031. Cet amendement vise ainsi à réintroduire ce à quoi nous tenons, et que je rappelle ici, à savoir un objectif intermédiaire commun,

Nous estimons que les territoires doivent pouvoir s’inscrire dans une dynamique commune, en suivant le même rythme. Le groupe socialiste est donc favorable à conserver une échéance nationale intermédiaire en 2035 et un objectif commun de réduction de moitié de la

En ce qui concerne l’amendement n° 165, et c’est tout le sens du dispositif que nous avons adopté en commission, nous considérons que la fixation d’un objectif chiffré au niveau national est trop rigide, et qu’il faut laisser à chaque région la possibilité de fixer son propre taux d’effort, en concertation avec les élus locaux représentés au sein de la conférence régionale

clair. Comme je l’ai indiqué en commission il y a quelques semaines, l’article 2, en supprimant l’objectif intermédiaire, n’incite pas les collectivités à faire évoluer leurs documents d’urbanisme sans attendre 2050.

Elles n’étaient donc pas en mesure de préparer l’évolution de leurs documents d’urbanisme ni d’assurer une maîtrise de leur consommation en cohérence avec des objectifs connus. Cela étant, la décennie de référence 2011 2021, au regard de laquelle l’effort de réduction doit s’apprécier, est maintenue,

au nom de la commission

Pour reprendre une citation cinématographique célèbre : « Le plus dur, ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage. » Voilà où réside l’hypocrisie de ce texte : si l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050 demeure,

vis à vis de leurs administrés, puisqu’ils conservent formellement leurs compétences urbanistiques, mais sont matériellement contraints par des régions, qui sont, comme je l’ai dit, très souvent hétérogènes.